ainsi que sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j’appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse

le Président de la République, puis votre ministre de l’économie ont dans le viseur les collectivités locales. Certains murmurent même déjà l’arrivée de contrats de Cahors de nouvelle génération

leurs agents. Elles ont dû s’y adapter malgré des budgets contraints, aux marges de manœuvre plus que restreintes quant aux recettes, à la différence de l’État. Monsieur le Premier ministre, quand cesserez vous de considérer les collectivités territoriales comme des supplétifs, face aux difficultés financières de l’État ?

d’abord, parce que je connais le très grand esprit de responsabilité des élus locaux et, ensuite, parce que nous sommes tous dans le même bateau. Quand on parle de la dépense publique, c’est bien la dépense de toutes les administrations publiques que l’on regarde.

L’Insee a dévoilé hier l’ampleur du déficit des finances publiques pour l’année 2023 : 5,5 % du PIB – c’est, selon les dires du Premier président de la Cour des comptes, un dérapage important et vraiment très rare.

le Premier président de la Cour des comptes, comme c’est l’usage, a présenté la conclusion du Haut Conseil des finances publiques (HCFP). On pouvait lire dans l’avis du 22 septembre 2023 Pour 2023, le Haut Conseil estime que les prévisions de prélèvements obligatoires du Gouvernement sont plausibles. » À mon sens, plutôt que de s’invectiver sur le sujet, mieux vaut comprendre… Assumer ! … comment l’inflation,

relataient l’histoire de Manon Dubois, Angevine de 23 ans, victime d’une soixantaine de faits d’agressions sexuelles reconnus par son agresseur comme par sa hiérarchie. Pourtant condamné par la justice, lui est toujours dans l’armée ; elle, elle n’y est plus, poussée à la démission par ses supérieurs. Selon votre ministère, la moitié des femmes militaires quittent nos armées avant la fin de leur carrière, alors même que la « grande muette » peine à recruter. Les problèmes d’agressions sexuelles ou racistes ne sont pas isolés, mais bien systémiques, comme le souligne la capitaine Saint Paul. Madame la secrétaire d’État, mes questions sont précises. Premièrement, la cellule Thémis ne compte que 4 agents pour 270 000 personnels : comptez vous la faire évoluer ? Deuxièmement, l’inscription au casier judiciaire n’empêche pas la poursuite de la carrière. Selon vous, est il possible qu’un agresseur reconnu demeure dans l’armée de la République ? Troisièmement et enfin, la Défenseure des droits

Il ne doit pas y avoir de tabou sur ce sujet, ni dans les armées ni ailleurs. M. le ministre l’a rappelé : porter l’uniforme de nos armées donne plus de devoirs que de droits. Néanmoins, dans les armées comme ailleurs, des dérives individuelles existent. Elles sont absolument inacceptables et il faut les traiter avec exemplarité. C’est pourquoi M. le ministre des armées a signé hier une instruction sur la conduite à tenir en cas de signalement.

Deuxièmement, sur les plans disciplinaire et judiciaire, le commandement doit être irréprochable. En cas de suspicion de viol ou d’agression sexuelle, des mesures de suspension conservatoire du mis en cause seront systématiquement prises lorsque les faits ont un caractère suffisant de vraisemblance. Aussi, une enquête disciplinaire doit systématiquement avoir lieu afin d’établir la matérialité des faits. Elle doit déboucher sur des sanctions disciplinaires de la plus grande sévérité. Troisièmement, que la victime présumée ait porté plainte ou non, le commandement doit systématiquement saisir le procureur de la République au titre de l’article 40

L’ensemble du Gouvernement est déterminé à agir pour lutter contre les violences faites aux femmes. Nous en faisons une priorité.

aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’une armée forte, à l’avant garde de la République et non logée en son arrière train. Dites le à nos généraux. Dites leur bien d’être rapidement dans le sens de l’Histoire s’ils veulent protéger l’institution

Les Républicains. Monsieur le garde des sceaux, pouvez vous me confirmer que, mardi dernier à Marseille, vous avez convoqué des magistrats du siège et du parquet que nous avions entendus dans le cadre de la commission d’enquête sur le narcotrafic, placée sous la présidence de notre collègue Jérôme Durain ? Pouvez vous confirmer que vous leur avez reproché d’avoir tenu le propos suivant : À Marseille, nous sommes en train de perdre la guerre contre le narcotrafic » ? Pouvez vous confirmer que vous leur avez reproché en tenant ces propos, fait prospérer le Rassemblement national ? Monsieur le garde des sceaux, pourquoi cette convocation ?

planification écologique, loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, plan de sobriété, stratégie nationale bas carbone ou encore plan d’investissement

C’est une très bonne nouvelle pour nos objectifs de décarbonation, que nous devons désormais amplifier. J’ajoute que cette baisse vaut

ministre délégué Frédéric Valletoux a rappelé dimanche dernier qu’une stratégie de déploiement des soins palliatifs avait été préparée, afin que les vingt et un départements qui n’en sont toujours pas dotés en bénéficient « avant la fin du débat sur la fin de vie tous ici ne pouvons que saluer une telle annonce. En effet, les équipes de soins palliatifs sont indispensables à la prise en charge de certains malades. accomplissent un travail extraordinaire, non seulement auprès des patients, mais aussi auprès des familles, qui se sentent parfois totalement démunies face à la situation de leur proche.

C’est absolument fondamental, car cette prise en charge est évidemment en lien étroit avec un éventuel souhait de recourir à l’aide à mourir. Nous ne pouvons donc qu’encourager le déploiement des services Madame la ministre, ma question est double. La première porte sur le calendrier. Je le répète, on nous a assuré que les départements seraient tous dotés de services de soins palliatifs avant la fin du débat sur la fin de vie

150 postes sont vacants dans l’ensemble des services existants et un quart des médecins vont quitter leurs fonctions d’ici à cinq ans. La parole

Madame la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, l’école, cette institution qui devrait être le symbole de l’égalité des chances, est aujourd’hui en proie à une crise sans précédent. Les enseignants, les parents d’élèves et les élus sont tous mobilisés depuis près d’un mois pour réclamer la mise en place d’un plan d’urgence pour l’éducation en Seine Saint Denis. Dans ce département, les classes sont surchargées, les enseignants sont épuisés, les locaux se dégradent, les professeurs ne sont pas remplacés. Face à cette situation, que fait le Gouvernement ? Il y répond par une réforme, le « choc des savoirs », qui va faire de l’école un lieu de tri et d’exclusion, et des économies budgétaires, dans un domaine dont il prétend faire une priorité. Comment peut on parler de priorité quand on réduit le budget de l’éducation Comment peut on parler de priorité quand on met en péril le recrutement des enseignants ? Comment peut on parler de priorité quand on propose une réforme qui risque de creuser les inégalités, d’affaiblir notre système éducatif et de compromettre l’avenir de nos enfants ? Nous luttons depuis près d’un mois pour que l’éducation soit considérée comme une priorité. Combien de fois devrons nous rappeler que l’éducation n’est pas un coût, mais un investissement : un investissement dans l’avenir de nos enfants, un investissement dans l’avenir de notre pays ? Combien de temps allons nous devoir encore nous battre pour que chaque enfant, quel que soit son lieu de résidence, ait accès à une éducation de qualité ? La Seine Saint Denis n’est pas le seul département concerné les syndicats d’enseignants appellent à la grève le mardi 2 avril, preuve que cette crise s’étend à l’échelle nationale ! Madame la ministre, quelle mesure concrète allez vous prendre pour mettre en place un plan d’urgence pour l’école publique en Seine Saint Denis ? Saint Denis ? Je vous demande également de bien vouloir recevoir une délégation de sénateurs de Seine Saint Denis qui, comme moi, sont préoccupés par l’avenir de nos enfants et croient en l’éducation, en son pouvoir de changer des vies, de transformer des sociétés et de construire un avenir meilleur. La parole

Une époque où, par la magie du 49.3, le Parlement peut au mieux soumettre ses propositions, sans pour autant peser en quoi que ce soit sur les équilibres budgétaires présentés par l’exécutif. Au moins pouvait on espérer que, en maîtrisant de bout en bout l’exercice budgétaire, le Gouvernement tiendrait les finances du pays, comme il s’y est engagé auprès des Français et de ses partenaires européens. Aujourd’hui, les faits sont là.

de la loi de programmation, afin de retrouver un peu de crédibilité internationale. Une époque formidable, disais je… Monsieur le ministre, vos coups de rabot n’ont aucun sens. Êtes vous prêt à rouvrir avec le Parlement le débat sur le budget dans son ensemble, tant sur les dépenses que sur les recettes ?

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, la rumeur qui bruissait depuis la semaine dernière a donc été confirmée par l’Insee ce mardi, dont les conclusions font froid dans le dos notre déficit public accuse une dégradation de 0,6 point par rapport à l’objectif que le Gouvernement s’était fixé, atteignant ainsi le creux vertigineux de 5,5 % du PIB pour 2024. Ces nouvelles prévisions placent la France parmi les pays aux finances publiques les plus dégradées de la zone euro, comme l’a indiqué la Cour des comptes dans son rapport annuel. Le Sénat avait pourtant tenté de marquer le pas lors de l’examen du projet de loi de finances. Il avait ainsi permis de dégager 7 milliards d’euros d’économies. Hélas ! parmi les nombreuses mesures que nous avions proposées, vous n’en avez retenu aucune

Monsieur le ministre, vous qui êtes amateur de littérature, et même auteur à vos heures perdues, je vous invite à méditer sur ces mots de Montaigne : « L’obstination et ardeur d’opinion est la plus sûre preuve de bêtise. » Le président du Sénat,

Cette politique constitue pourtant le cadre fondamental de l’action à mener pour toutes les filières françaises et concerne tous les Français dans leur vie quotidienne. Elle est, en définitive, la carte et la boussole dont la France se dote pour atteindre les objectifs climatiques et environnementaux pris dans les cadres européen et mondial.

comment faites vous face à ces obligations et à leur financement dans un contexte de dégradation accrue des finances publiques, de dynamique économique atone et de difficultés sociales particulièrement préoccupantes ?

vous chantiez les louanges d’un monde nouveau. Sept ans plus tard, vous tournez le dos à l’ambition d’une France résiliente et solidaire pour le monde de demain. Pis encore, vous poursuivez méthodiquement le saccage de l’État providence, alors que rien d’efficace ne se fera sans justice sociale.

des outre mer, à Orléans, la rumeur enfle selon laquelle des sans domicile fixe (SDF), dont beaucoup de migrants, seraient déplacés en province pour faire place nette à Paris en prévision des jeux Olympiques. Ces SDF partiraient régulièrement à bord de bus à destination de Strasbourg, d’Angers et d’Orléans – et sans doute d’autres villes. Malgré ses demandes répétées auprès de l’État, le maire d’Orléans n’obtient que des réponses évasives. Il est inacceptable qu’un maire apprenne de telles informations par voie de presse de presse ! Le Gouvernement prétend vouloir instaurer des relations de confiance avec les collectivités. Aussi, il est temps d’accorder un minimum de considération aux élus locaux et de les tenir informés de ce type d’opérations., ce sont, comme toujours, les maires qui devront trouver des solutions.

pour les riverains parisiens. Cette politique de façade, les villes de province n’en veulent pas, pas plus qu’elles ne souhaitent être les victimes d’une politique migratoire défaillante

des outre mer. Alors que la France s’apprête à accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, un événement d’une ampleur inégalée qui marquera l’histoire de notre pays, une question de sécurité cruciale se pose. Avec la mobilisation exceptionnelle annoncée de 30 000 policiers et gendarmes chaque jour pour garantir la sécurité de cet événement, notamment à Paris et en Seine Saint Denis, on ne peut que se féliciter de l’ampleur des dispositifs prévus pour faire face aux diverses menaces, qu’elles soient terroristes ou d’ordre public. En témoigne le passage récent au niveau « urgence attentat Cette mobilisation sans précédent, équivalant à une opération de sécurité que la France n’a jamais mise en place – selon vos dires, monsieur le ministre –, suscite néanmoins une préoccupation majeure pour les territoires en dehors de la capitale. Le repositionnement stratégique des forces de l’ordre, incluant la fin de la distinction entre zones de police et de gendarmerie pour la durée des jeux, permettra certes une flexibilité opérationnelle accrue, mais pose la question de l’impact sur la sécurité des villes de province. Ces dernières, en fournissant une part significative de leurs effectifs à la capitale, pourraient se retrouver dans une situation de vulnérabilité face à des événements de criminalité, tels que des émeutes urbaines. Dans ce contexte, quelles mesures quelles mesures le Gouvernement envisage t il de mettre en œuvre pour assurer que la sécurité des villes de province ne soit pas compromise par cette redistribution des forces de l’ordre ? Comment garantir que la sécurité de l’ensemble du territoire reste une priorité, sans créer de déséquilibre préjudiciable à la tranquillité publique et à la réponse aux urgences locales ? La parole

Or Coallia vient de faire l’objet d’un rapport édifiant de la Cour des comptes, lequel fait apparaître que cette association, confrontée à toujours plus de sollicitations de l’État pour répondre aux besoins en hébergement d’urgence, eux mêmes sans cesse croissants en raison de la pression migratoire, est dans une situation très préoccupante. En 2017, elle a frôlé le dépôt de bilan. Depuis lors, la Cour des comptes observe que Coallia ne maîtrise pas sa croissance due aux sollicitations grandissantes de l’État. Pis encore, l’association avoue ne plus savoir qui elle accueille dans ses centres et, plus précisément, dans quelles conditions : aucune procédure n’existe pour faire remonter d’éventuels événements graves. La Cour des comptes en conclut qu’il est urgent pour l’État de se préoccuper de l’avenir de Coallia,

Quand comptez vous exercer votre contrôle sur les différentes associations subventionnées à un niveau exceptionnellement élevé et intervenant dans le domaine de l’immigration ? N’est il pas temps de mettre un terme à cette fuite en avant dans laquelle l’État, dépassé par une pression migratoire dont il a pourtant l’entière s’en remet par facilité à des associations ? Celles ci y répondent en effet tant bien que mal, voire de manière préoccupante, au coup par coup, dans l’indifférence évidente de leur donneur d’ordre et principal bailleur de fonds : l’État.

quelle est votre vision de la souveraineté industrielle de notre pays ?

ont mis en place la recherche d’un repreneur. Ils ont décidé la semaine dernière de se mettre sous la protection des procédures collectives pour accélérer ce processus. Sur ce dossier, comme sur tous les autres, monsieur le sénateur, je vais agir de la même manière

Les PFAS sont partout, et dans mon département, l’Isère, comme chez mes voisins du Rhône, de la Loire et à de nombreux endroits en France, les alertes se multiplient sur la qualité des eaux de consommation. Les maires se trouvent démunis, ainsi que les services de l’État, je le Monsieur le ministre, la mise en place d’un plan d’action pour prévenir les rejets de PFAS, en bonne intelligence avec nos industriels, est une bonne chose, mais ce plan ne traite que le problème en amont, car pour l’aval, il est trop tard. Pour nos territoires, il n’est plus temps de se demander comment réduire ces polluants : il faut les détruire.

contrairement à ce que certains activistes tentent de faire croire, l’autoroute Castres Toulouse n’est pas un projet, mais bel et bien une réalité : elle est déjà à moitié achevée. Chaque jour, plus de 800 ouvriers, compagnons et ingénieurs travaillent d’arrache pied pour la réalisation de cette artère vitale tant attendue par toutes les forces vives du sud du Tarn. Les opposants, de moins en moins nombreux, venant de plus en plus loin et de plus en plus radicalisés, ont perdu tous les recours devant la justice administrative ; nombre d’entre eux ont été lourdement condamnés pour violences par la justice pénale. Ils essaient encore, au travers de sabotages d’occupations illégales d’arbres, de faire diversion et de retarder le chantier. Quelle n’a pas été notre surprise de voir l’ONU, par le biais d’un pseudo expert rapporteur, prendre position sur le maintien de l’ordre autour de ce chantier légal,

totalement scandaleuses, uniquement à charge et élaborées sans que les défenseurs du projet, acteurs économiques, élus locaux et parlementaires, aient été auditionnés, nous interpellent. Alors que la France est l’un des principaux contributeurs des Nations unies et qu’elle est un État de droit, une démocratie, quelle est la position du Gouvernement sur ce rapport ?

Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin. L’ordre du jour appelle l’examen de la demande de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête afin de mener une mission d’information relative à l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors des séances des 19 et 26 mars

pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour mener cette mission d’information. Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient

pénitentiaire (DAP) souhaite en effet bénéficier du dispositif d’affectation des biens meubles saisis dans le cadre des enquêtes de police, notamment des drones qui sont utilisés pour effectuer des livraisons illicites en détention.

situation, cet amendement vise à rendre obligatoire, sauf motivation contraire, la confiscation des biens meubles ou immeubles dont l’origine n’a pu être justifiée, en cas de délit ou de crime puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect à leur auteur.

qu’au moment même où nous convenons tous que la confiscation des avoirs criminels demeure la matrice d’une lutte efficace, ces amendements visent à combler un vide juridique et à faciliter le travail de la justice. Celui ci est essentiel à la mise en place d’un système qui sanctionne effectivement les montages financiers

propriétaire d’un commerce ou détenant des participations dans diverses sociétés acquis avec de l’argent sale et disposant d’autres biens, a aujourd’hui la possibilité de conserver tous ces biens et de continuer à en disposer. tend par ailleurs à modifier le cinquième alinéa de l’article 1 afin de combler un vide juridique en ce qui concerne la confiscation des biens meubles ou immeubles dans les cas où le condamné n’a pu en justifier Au demeurant, ce dispositif répond aux préconisations de l’article 5 de la directive 2014 42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.

également que le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement peuvent refuser la restitution d’un bien saisi constituant l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction en l’absence de condamnation pénale.

n° 11 rectifié.

des biens confisqués. Nous en sommes convaincus, l’État doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leur sont rendus, et que le crime organisé ne l’emporte pas sur la défense du bien commun. Quel est l’avis de la commission

en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l’éducation à la citoyenneté par l’éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Il paraît donc de bon sens d’ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués. Cela contribuera à renforcer l’économie sociale et solidaire et l’entreprenariat social, tout en luttant contre le crime organisé.

M. Ian Brossat. Cet amendement vise à élargir le conseil d’administration de l’Agrasc en y incluant des représentants du Parlement, des associations de victimes et des organismes dont l’objet est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou encore la défense des personnes en situation d’expulsion. Il s’agit en effet d’améliorer les pratiques de mise à disposition des biens confisqués.

Ces nominations renforceraient la capacité d’action de l’Agence en faveur du monde de l’entrepreneuriat social et du logement pour les plus démunis. très bien défendu.

entraîne une privation du droit de propriété. Il faut donc prévoir que puisse être contestée devant une juridiction la privation du droit de propriété portant sur un bien saisi. Pour cela, il est essentiel qu’un tel recours présente à la fois un caractère contradictoire et suspensif ; sinon, nous craignons que le dispositif ne soit censuré par le Conseil constitutionnel.

le code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit à la partie civile en matière de saisie spéciale. Tel est

de s’en prendre aux biens de la délinquance : on commence par les saisir, c’est à dire par les rendre indisponibles juridiquement, et l’on finit par les confisquer, c’est à dire par transférer leurs droits de propriété à l’État.

M. Ian Brossat. Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée à l’Assemblée nationale et supprimée en commission. Celle ci a pour objet d’encourager la formation des magistrats et des services de police judiciaire sur la question des saisies et des confiscations des avoirs criminels. Quel est l’avis de la commission

vous l’avez compris, la saisie des biens intervient au stade de l’enquête, tout comme la décision de leur affectation. Toutefois, dès lors que la juridiction de jugement est saisie, il n’existe plus de procédure qui puisse permettre, par exemple, de vendre un bien dont il serait justifié de se dessaisir. C’est pourquoi je vous propose, par cet amendement –

Je préfère le maintien de la compétence du Parquet ou du juge des libertés et de la détention (JLD), car elle est plus simple en pratique s’agissant de l’exercice d’une compétence qui n’est subordonnée à aucune demande du propriétaire. En effet, il est illusoire d’envisager qu’un président de cour d’assises se penchera sur un dossier, en amont de l’audience, pour prendre l’initiative sur une décision d’affectation ou de vente des biens meubles saisis dans le cadre de l’information judiciaire.

constitutionnelles en matière d’atteinte au droit de propriété et au droit à un procès équitable. Je l’ai déjà dit précédemment, mais je n’ai pas été convaincant – sans doute n’ai je pas trouvé les bons mots. Toutefois, je persiste à vous dire que je suis, bien évidemment, défavorable à cet amendement.

Cela permettra de renforcer l’efficacité de notre arsenal pénal en la matière, tout en maintenant les équilibres fondamentaux de notre droit, qui suppose qu’une telle peine soit justifiée, adaptée et proportionnée.

Cet amendement vise à permettre le prononcé d’une peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine

portant sur le sort des biens saisis, à compter de la saisine de la juridiction de jugement et tant qu’elle n’a pas statué au fond. Il s’agit de clarifier les règles de compétence applicables au contentieux des saisies à ce stade de la procédure. Quel est l’avis de la commission ? Par cet

» concernait également les titulaires de baux et qu’il fallait protéger ceux qui étaient de bonne foi. C’est pourquoi, en commission, nous avons fait admettre que l’expulsion ne devait pas viser les titulaires de baux avant la saisie. L’avis est donc défavorable sur cet amendement, qui est contraire à ce qui a été voté en commission. l’amendement précisent que la décision de confiscation d’un immeuble ne vaut pas titre d’expulsion à l’égard de tous les titulaires d’un bail. J’ai cru comprendre que vous étiez d’accord avec

la notion de biens mal acquis désigne des avoirs ou des biens ayant été détournés du budget d’une organisation internationale, d’un État ou d’une entreprise publique pour une personnalité politiquement exposée et placés à l’étranger à des fins personnelles.

politiquement exposées, et non plus seulement par celles qui exercent des fonctions publiques dans l’État concerné. Je rappelle que le mécanisme de restitution des biens mal acquis, créé par la loi du 4 août 2021,

Actuellement, le dispositif est applicable aux infractions commises par « une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat

La séance est reprise. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous arrivons au terme de la procédure d’examen parlementaire du projet de loi

nationale, car il est au cœur de l’insertion sociale et économique de nos concitoyens. Sans logement, point de vie dans nos villes et dans nos villages

des dispositifs introduits par le Sénat. Nous souhaitions renforcer les outils à disposition des maires pour traiter les petites copropriétés dégradées.

adaptée à celle de l’opération. Le maire en fixera la date de fin et elles pourront être renouvelées en fonction du besoin.

vous retrouverez également dans ce texte les mesures pour faciliter la réalisation des travaux et la gestion des copropriétés auxquelles nous étions attachés. a consacré la création d’un nouveau prêt global et collectif aux copropriétés et a tenu compte de notre préoccupation de faire en sorte que les banques et les cautions s’y engagent véritablement. Pour cela, il fallait que la copropriété ne soit pas une boîte noire financière. Ainsi, les prêteurs et les organismes de garantie pourront donc consulter le fichier de la Banque de France des incidents de paiement et obtenir du syndic des informations complètes pour acquérir une juste vision du risque et de l’état de la copropriété.

En matière de lutte contre les marchands de sommeil, nos deux assemblées se sont accordées pour alourdir les peines d’amende et de prison, et pour interdire à ces derniers d’acquérir un bien immobilier dans un cadre juridique

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux de me retrouver devant vous aujourd’hui, un mois jour pour jour après avoir eu l’honneur de défendre ici le projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce beau texte. Je tiens à saluer l’apport des sénateurs, et tout particulièrement l’engagement et le travail de la rapporteure Amel Gacquerre et de la présidente de la commission Dominique Estrosi Sassone, avec qui nous avons eu des échanges nourris et constructifs tout au long de l’examen Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à l’ensemble des partis politiques qui se sont particulièrement investis sur ce texte pour assurer son adoption par le Sénat en première lecture à l’unanimité des votants, comme l’a rappelé Mme la rapporteure. a été l’occasion, grâce aux efforts des parlementaires des deux assemblées, de sécuriser, d’enrichir et d’améliorer les dispositions d’un projet de loi utile et nécessaire. Je formule le vœu de retrouver ce même esprit de construction sur les textes que nous aurons à étudier à l’avenir. En effet, la version du texte qui vous est soumise aujourd’hui est le fruit d’un travail parlementaire ambitieux.

pays. Sur ce sujet, mesdames, messieurs les sénateurs, nous partageons le même diagnostic et le même constat : il est tout simplement intolérable que des personnes continuent de vivre dans notre pays dans des conditions d’habitat dégradé, indécent ou indigne.

d’abord, nous aidons les copropriétés à emprunter les sommes nécessaires pour réaliser les travaux de rénovation. Ensuite, nous renforçons les outils à disposition des élus et des opérateurs pour mener de grands projets de réhabilitation. Enfin, nous augmentons les sanctions contre ceux qui tirent profit de la dégradation de l’habitat.

Mathieu Hanotin, maire socialiste de Saint Denis, et Michèle Lutz, maire Les Républicains de Mulhouse, pour explorer les moyens d’améliorer la prise en charge de ces situations difficiles. Leurs travaux ont permis à mon prédécesseur Patrice Vergriete d’élaborer le texte à la fois pragmatique et ambitieux qui vous a été soumis. Pour Pour mieux traiter les situations de dégradation de l’habitat, il nous faut mieux les anticiper. Ces processus mettant plusieurs années à s’installer, ils doivent être traités plus en amont. Dans notre vie comme dans celle des bâtiments, il vaut toujours mieux agir avant qu’il ne soit trop tard. Avec ce texte, notre philosophie est simple : mieux vaut prévenir que guérir ou détruire. Dans cette optique, le projet de loi crée notamment, à l’article 3, une nouvelle procédure d’expropriation, qui permettra d’intervenir plus en amont du cycle de dégradation des copropriétés. Je me réjouis que les travaux de nos rapporteurs aient permis de conserver des apports ambitieux à cet article 2, qui était particulièrement attendu, permettra aux syndicats de copropriété d’assurer le financement des travaux au moyen d’un emprunt collectif. Il s’agit d’une innovation majeure, qui fera gagner plusieurs mois d’examen de dossiers individuels, au profit d’une approche collective et globale. le temps est un allié précieux pour éviter une dégradation trop profonde des copropriétés. La rédaction adoptée en commission mixte paritaire constitue un compromis salutaire entre les positions des deux chambres, qui permettra aux copropriétés d’emprunter

de ce texte, nous poursuivons également la lutte que nous avons engagée dès 2017 contre les marchands de sommeil. Je le rappelle avec fermeté : dans notre pays, nul n’a le droit de tirer une rente de la vulnérabilité d’autrui. Sur l’initiative des parlementaires,

Cet article permettra, dans le cadre de projets partenariaux d’aménagement (PPA) et d’opérations d’intérêt national (OIN), de débloquer rapidement les procédures liées aux exigences environnementales et urbanistiques afin de gagner plusieurs mois précieux lors du lancement d’un projet.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en adoptant ce projet de loi, nous nous doterons de nouvelles capacités pour lutter contre l’habitat indigne, et ce de manière pragmatique, opérationnelle et transpartisane. Au travers de ce texte, nous nous attaquons à la question des copropriétés dégradées en ayant un objectif précis en tête

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte,

Il aurait été plus réjouissant encore que, à côté de l’accélération et de la simplification, le Gouvernement ajoute un volet financement qui aurait permis d’aller plus loin en vue de véritablement résoudre la situation des occupants des plus de 1,5 million de logements relevant d’une copropriété en difficulté.

Tous types de logements confondus, plus de 12 millions de personnes sont fragilisées par la crise du logement. Il s’agit d’une véritable bombe sociale. Le montant total des travaux nécessaires pour rénover l’habitat dégradé, prévenir la fragilisation de nouvelles copropriétés et tenir les objectifs de rénovation énergétique serait d’au moins 9 milliards d’euros. Cette somme paraît inaccessible sans intervention publique, dans un contexte d’inflation galopante et de perte de pouvoir d’achat qui n’épargne personne au sein des classes moyennes et populaires, ni les propriétaires ni les locataires. Les procédures sont simplifiées, mais quelle collectivité aura les moyens de les déclencher ? Des prêts collectifs sont créés, mais quelle copropriété aura les moyens d’emprunter ? Pour les collectivités, nous facilitons les interventions des agents assermentés et étendons la possibilité de recourir au permis de louer, mais où sont les agents publics qui mèneront à bien ces nouvelles missions ? Nous facilitons les expropriations, mais comment assurerons nous le paiement exigé par la loi ? L’obligation de résultat qui incombe aux administrations publiques est confrontée aux coupes budgétaires imposées par le Gouvernement. Comme d’autres avant elle, à défaut de financement, cette loi restera une bétonnière qui attend son ciment.

Ces situations insupportables pour celles et pour ceux qui vivent dans un logement indigne ou dans une copropriété dégradée ne doivent laisser personne indifférent. Pour notre part, nous soutenons les 2,4 millions de demandeurs d’un logement social qui attendent une réponse positive. Nous soutenons les locataires qui paient des loyers exorbitants dans le parc privé et qui sacrifient d’autres dépenses pour éviter l’expulsion, que le Gouvernement et la majorité sénatoriale ont facilitée. De même, nous soutenons particulièrement les propriétaires occupants, dont 200 000 vivent dans une copropriété dégradée.

Ce n’est d’ailleurs pas en révisant les critères du diagnostic de performance énergétique afin de remettre 140 000 passoires thermiques sur le marché locatif que l’on résoudra une crise dont les fondations sont aussi complexes que multifactorielles.

40 % des Français habitaient dans un immeuble collectif. La qualité de cet habitat doit donc devenir une priorité de notre action politique, puisque l’habitat dégradé est un phénomène silencieux et massif encore largement méconnu, qui ne concerne pas seulement quelques villes pauvres ou quelques quartiers prioritaires. Il s’agit non seulement d’un stock de logements à réhabiliter, mais d’un flux qui se renouvelle : de nouveaux logements se dégradent tout en restant habités, parce que d’autres logements abordables manquent et que les personnes exclues sont toujours plus nombreuses. Pourtant,

Certes, ce texte n’a pas la prétention de résoudre toutes les causes de la crise du secteur du logement. Reconnaissons toutefois qu’il apporte sa pierre à l’édifice de deux chantiers titanesques, la rénovation de l’habitat dégradé et les grandes opérations d’aménagement.

Concrètement, les élus pourront agir en cas d’urgence, par exemple « si les travaux entrepris […] ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé

Trop de nos concitoyens subissent des désagréments liés à l’immobilisme des uns ou à l’irresponsabilité des autres. Les maires pourront également s’appuyer sur un rapport du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) pour motiver leurs arrêtés de mise en sécurité. le préfet ou leurs représentants pourront également participer à l’assemblée générale d’une copropriété, étape qui permet bien souvent de recenser les premiers signes de la dégradation du bâti. bâti. Ces mesures utiles permettent de donner plus d’outils aux acteurs de terrains, qui restent les plus compétents pour prendre ces décisions. Ensuite, mes chers collègues, si nous voulons accélérer et faciliter la rénovation

De plus, il faut bien admettre que les copropriétaires demandent davantage d’accompagnement, notamment en matière de rénovation énergétique. Comme de tels travaux sont en général très onéreux, ils nécessitent la plupart du temps l’octroi d’un prêt.

Encore une fois, l’objectif est clair : avoir une vision complète des capacités financières de la copropriété pour s’assurer de sa pérennité. Enfin, mes chers collègues, au delà des objectifs de simplification et d’accélération, l’adoption de ce texte permettra également de renforcer notre lutte contre un fléau qui gâche le quotidien de nombreux Français : celui des marchands de sommeil.

produit. Parce que nous accordons de nouvelles attributions aux élus locaux, parce que nous accompagnons les copropriétaires dans leurs travaux de rénovation, parce que nous renforçons la lutte contre les marchands de sommeil, nous parviendrons bel et bien avec ce projet de loi à simplifier la rénovation des copropriétés dégradées et à accélérer les grandes opérations d’aménagement.

est une bonne loi, nécessaire. Il traduit le besoin d’adapter les outils permettant à la puissance publique et aux maires des villes concernées de lutter contre le phénomène de l’habitat indigne, véritable fléau qui gangrène des immeubles et des quartiers. Nous saluons le travail préparatoire réalisé par Mathieu Hanotin et Michèle Lutz : leurs propositions nous ont accompagnés efficacement dans le cadre de l’examen de ce texte. La majeure partie de nos suggestions ont été entendues en commission et en séance publique. À cet égard,

lors de la commission mixte paritaire, nous sommes satisfaits du compromis trouvé sur les colocations à baux multiples. En effet, les élus pourront refuser le permis de louer lorsqu’il apparaît que les locaux ne permettent pas d’assurer aux habitants des conditions de vie digne. Nous avons obtenu une avancée majeure concernant la prévention de l’habitat dégradé, y compris dans le bâti ancien, en permettant aux maires de demander la réalisation d’un diagnostic structurel. Historique ! Nous sommes très satisfaits que les discussions aient abouti sur ce point, car ces centres historiques, qui ne présentent pas toujours de signes extérieurs de dégradation, nécessitent une vigilance accrue et un outil permettant de détecter ce qui demeure souvent invisible. Enfin, à l’article 18, nous sommes particulièrement satisfaits

en matière d’habitat indigne dans les communes volontaires des six territoires d’accélération. En ce qui concerne l’installation d’hébergement d’urgence, j’ai rappelé notre opposition non pas au recours à des bâtiments modulaires et déplaçables, mais à la dispense de toute règle d’urbanisme.

que j’ai rappelées, nous voterons en faveur des conclusions de cette commission mixte paritaire. Toutefois, rappelons que face à une crise du logement qui s’aggrave, sortir de l’habitat indigne impose aussi de disposer d’une offre de logements adaptés aux revenus et aux besoins des Français. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demande donc un moratoire je vous remercie

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis qu’après le travail approfondi de nos rapporteurs, les deux assemblées se soient entendues pour marquer leur détermination à lutter contre l’habitat dégradé.

Contrairement à bien des textes qui viennent des bureaux parisiens, cette loi vient des demandes des maires et des remontées du terrain. En examinant ce projet de loi, la commission des affaires économiques du Sénat a voulu renforcer son caractère pragmatique et opérationnel.

nous avons aussi consulté les maires sur la plateforme internet du Sénat pour mieux comprendre leurs attentes, leurs aspirations et leurs besoins.

ou encore celles relatives au contrôle structurel des bâtiments, inspirées de Mulhouse ou de Lille. Je suis également satisfaite que nous ayons pu éviter de tomber dans le syndic .

les syndics ont plus besoin d’être confortés dans leurs missions que d’être jetés en pâture d’une éventuelle dérégulation. Justement, en matière de simplification, ce projet de loi permettra de développer l’usage du numérique entre les syndics et les copropriétaires.

Face à la crise, nous aurons la responsabilité de voter des mesures ambitieuses et efficaces pour donner un logement à l’ensemble des Français et pour rééquilibrer le marché locatif.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’habitat dégradé et plus largement le logement constituent des problématiques parmi les plus préoccupantes dans notre pays. dégradé désigne généralement des conditions de logement en dessous des normes de salubrité, de sécurité et de décence requises. Ces situations se manifestent souvent dans les quartiers urbains défavorisés, transformés en ghettos, entraînant à tout le moins un sentiment d’insécurité, ainsi que l’augmentation des actes de délinquance et de violences. Dans ces environnements, les logements peuvent présenter diverses formes de dégradation, qui vont de l’insalubrité et de l’insécurité des structures aux problèmes d’humidité, de surpopulation et d’infestations parasitaires. Les multiples conséquences de l’habitat dégradé touchent tous les aspects de la vie quotidienne des habitants.

Du point de vue économique, l’habitat dégradé a un impact négatif sur la valeur immobilière des zones environnantes, ce qui peut entraîner un déclin économique et une désertification commerciale. De plus, les quartiers comprenant des logements insalubres se trouvent dans de grandes villes où les prix de l’immobilier explosent. Les étudiants et les familles précaires se retrouvent contraints de vivre dans ces logements. résoudre cette problématique complexe, tout le monde doit engager des efforts concertés pour améliorer les conditions de logement des populations affectées. Cela implique de mettre en œuvre des politiques publiques visant à garantir l’accès à un logement décent pour tous, ainsi que d’intégrer dans des programmes de rénovation urbaine des mesures de développement social et

Une réforme complète du système est attendue. Ce texte n’est qu’une étape, qui ne peut rester la seule. Nous devrons poursuivre nos efforts pour ajuster et moderniser nos outils. Encore une fois,

chers collègues, nous partageons bien entendu l’esprit de simplification et d’accélération de ce projet de loi, qui a pour but de prévenir et d’éviter le pire. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire nous semble équilibré. Le groupe Les Indépendants votera, bien entendu, en sa faveur. Très bien ! La parole

Je tiens de nouveau à remercier la rapporteure du texte, notre chère collègue Amel Gacquerre, qui a réalisé un travail impressionnant et salué par tous sur ces travées.

Par ailleurs, pour anticiper, prévenir et résoudre les problèmes rencontrés, les pouvoirs publics et les syndics doivent plus que jamais travailler de concert lorsque les propriétaires font défaut. Le chapitre II prévoit des mesures pour accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés. Ainsi, les pouvoirs du maire se trouvent renforcés par la sécurisation du cadre juridique relatif aux expropriations, qui était à la sécurité des citoyens et indispensable au recyclage des habitats urbains. Il en est de même quant à l’application des mesures de démolition des constructions jugées irrégulières ou présentant des risques pour la sécurité et la santé des résidents. Ce texte est un premier pas, et pour cette raison nous adopterons les conclusions de la commission mixte paritaire. Mais la suite reste à écrire : il faut désormais accompagner nos maires pour qu’ils s’approprient les outils législatifs, débloquer les moyens nécessaires et faciliter l’accès aux aides à l’investissement. Le Gouvernement avait promis des mesures structurantes, et je ne peux que regretter la portée restreinte de ce texte. Monsieur le ministre, la décentralisation annoncée ne suffira pas.

amender et améliorer la loi SRU est une bonne chose, poursuivre la simplification également, mais il nous faut des mesures fortes, à la hauteur de la situation. Nous connaissons votre feuille de route et nous voyons votre bonne volonté. Vous avez lancé, pas plus tard qu’hier, une mission en faveur du choc d’offre par le soutien à l’investissement, mais nous attendons plus de mesures concrètes. Ne soyons pas effrayés ou intimidés devant l’immensité de la tâche : ayons le courage de mener ce combat, d’engager les moyens nécessaires et d’avoir une politique ambitieuse pour le logement de demain

dans la lutte contre l’habitat dégradé et dans la protection des occupants vulnérables. Il répond aux attentes des acteurs de terrain, notamment des élus locaux ; d’ailleurs, il s’est inspiré du rapport de Michèle Lutz et de Mathieu Hanotin, qui est présent dans notre tribune

des avancées que je tiens à souligner. Je pense par exemple au renforcement des moyens de lutte et de sanctions pénales contre les marchands de sommeil, à sommeil, à l’élargissement de la couverture assurée par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l’extension du champ d’intervention de l’association Foncière Logement ou encore à la facilitation des travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés, grâce au passage de la règle de l’unanimité à celle de la majorité absolue.

aussi un très net recul. Une fois de plus, nous avons cédé au lobby des syndics, et ma voisine de 88 ans ne vous remercie pas… Vous l’aurez compris, pour les écologistes, si ce texte va globalement dans la bonne direction, il reste des loupés. me réjouis néanmoins que nous poursuivions le travail et les auditions dans le cadre de la commission d’enquête sur la paupérisation des copropriétés, demandée par nos amis communistes.

Les droits des locataires sont bafoués, sacrifiés sur l’autel de la rentabilité du meublé touristique pour les quelques semaines des Jeux. C’est une pratique illégale et c’est surtout une catastrophe pour le logement de nos concitoyens parisiens ou grands parisiens. Je salue d’ailleurs l’initiative de notre collègue sénateur de Paris, Ian Brossat, qui a déposé une proposition de loi visant à instaurer une trêve olympique des expulsions locatives. Il faut agir en faveur du logement, monsieur le ministre, et il faut même accélérer. L’accès à un logement digne, à un logement durable, devient de plus en plus difficile. Pour les écologistes, le logement ne doit pas être un produit financier au bénéfice des 10 % des Français les plus riches, qui détiennent 44

J’ajoute que la suppression de 2,14 milliards d’euros d’autorisations d’engagement consacrées au dispositif MaPrimeRénov’ est incompréhensible. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour ne pas vous laisser corseter par Bercy… Pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour répondre à la crise du logement en France. Nous voterons ce texte, mais il est essentiel que celui ci soit soutenu par des ressources et des compétences, notamment pour les petites collectivités, et nous attendons fermement des mesures ambitieuses

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie

la commission mixte paritaire préserve, pour l’essentiel, l’équilibre du texte adopté par le Sénat, qui avait veillé à recentrer la proposition de loi sur les mesures susceptibles d’avoir un impact réel et positif. égard aux enjeux liés au vieillissement de la population et aux besoins considérables qui s’annoncent, cette proposition de loi fait figure de texte d’attente. Le vote dans les mêmes termes par les deux assemblées de l’article 2 B souligne l’impérieuse nécessité de mettre rapidement à l’ordre du jour un projet de loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, afin de donner aux acteurs, aux professionnels et aux usagers une lisibilité concrète sur les moyens qui seront mis en œuvre pour une politique de l’autonomie à la hauteur des enjeux. Il est particulièrement urgent de prendre à bras le corps le sujet de l’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie, notamment ceux de l’aide et de l’accompagnement à domicile, si l’on veut réussir le « virage domiciliaire ». Cela passe notamment par la revalorisation de la rémunération de ces professionnels, mais d’autres leviers devront être actionnés, comme la création d’une spécialisation en gériatrie de l’exercice infirmier en pratique avancée, que j’appelle de mes vœux. Le texte que nous examinons sans doute pour la dernière fois aujourd’hui contient cependant certaines avancées qui justifient de le soutenir. d’abord, la création du service public départemental de l’autonomie (SPDA) vise un double objectif de décloisonnement des politiques sanitaires et médico sociales et de rapprochement des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. mixte paritaire conserve les principaux apports des deux assemblées. Le dispositif proposé présente l’avantage de la souplesse et de l’adaptabilité aux réalités locales, car la réponse aux objectifs du SPDA pourra varier selon les territoires. Le texte confirme l’inscription territoriale du SPDA, qui sera l’instance de coordination et de planification pluriannuelle des politiques de l’autonomie. La réintroduction à l’article 1 de la conférence nationale de l’autonomie, dans un format moins institutionnel, sur le modèle de la Conférence nationale du handicap, permettra de donner une impulsion à la politique de prévention de la perte d’autonomie sans créer de structure complexifiant le paysage. Je considère que la logique de parcours doit être un pilier du SPDA, lequel doit s’inscrire dans la perspective du virage domiciliaire et favoriser un continuum des modes d’accompagnement et de soins. Ceux ci incluent naturellement le maintien à domicile, qui devra être rendu possible dès lors qu’il correspondra au souhait de la personne âgée, mais aussi l’habitat intermédiaire – résidences autonomie, résidences services, habitat inclusif (Ehpad), qui reste nécessaire et dont la place doit être repensée et mieux valorisée, ainsi que, dans certains cas, l’hospitalisation en unité de soins de longue durée. La coopération au sein de groupements, que le texte encourage et rend obligatoire pour les établissements et services publics autonomes, et la prise en compte dans ce cadre des personnes en situation de handicap vieillissantes participent également de cette logique de parcours. paritaire est revenue sur la disposition prévoyant un avis du président du conseil départemental sur la nomination des directeurs d’Ehpad publics, considérant qu’elle aurait remis en cause la répartition des compétences avec les maires. Le développement de la prévention de la perte d’autonomie constitue un autre axe structurant du texte. Dans cette perspective, la généralisation du programme Icope (, ou soins intégrés aux personnes Conformément à la rédaction du Sénat, le texte clarifie l’articulation de ce programme avec le dispositif des rendez vous de prévention. Pour ce qui concerne le volet du texte relatif aux conditions d’accueil et de prise en charge des résidents en Ehpad, la commission mixte paritaire n’a retenu que les dispositions apportant de réelles améliorations pour les usagers. également confirmé la création d’un droit pour les résidents d’Ehpad d’accueillir leur animal domestique au sein des établissements, en prenant en compte la volonté du Sénat d’encadrer ce droit pour garantir la santé et la sécurité des résidents et du personnel, ainsi ainsi que le bien être des animaux. Un arrêté précisera donc les catégories d’animaux domestiques pouvant être accueillis et les conditions d’hygiène et de sécurité qui devront être respectées. Introduite par le Sénat, la possibilité ouverte aux Ehpad dont la capacité d’accueil est intérieure à un seuil fixé par décret d’offrir des places d’accueil de jour sans se voir opposer le plancher existant de places offertes a été confirmée par la commission mixte paritaire dans une rédaction de compromis. En outre, l’accueil de jour

qui étaient déjà satisfaits ou qui n’apportaient pas d’améliorations significatives aux prérogatives de contrôle, déjà robustes et récemment renforcées à la suite du scandale Orpea. La qualité et la sécurité de la prise en charge passent dorénavant par l’allocation des moyens nécessaires au contrôle de l’ensemble des établissements dans la durée. Ainsi, même s’il ne constitue qu’une étape et n’est nullement un aboutissement, je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte

la transition démographique nous conduit d’ici à 2030 vers une société où les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Ce qui est devant nous, c’est une société au visage nouveau une société de la longévité. Oui, nous vivons plus longtemps, et cela nous impose de tracer ensemble le cap d’une société préparée à cet immense défi. C’est à cette seule condition que la transition démographique sera une chance pour tous et non un fardeau. En ce sens, le chantier du grand âge est essentiel, je dirais même existentiel, pour notre pays. J’ai d’emblée évoqué ce sujet comme une question de société qui nous concerne tous, car, au delà des questions de santé publique et des enjeux évidents de prise en charge de la perte d’autonomie posés par le vieillissement de notre population, les rapports que nous entretenons collectivement avec nos aînés disent beaucoup de l’état d’une société. En France, la solidarité entre les générations est le fondement même de notre modèle de protection sociale et même, plus généralement, de notre contrat social. C’est quelque chose dont il faut être fier, qu’il faut préserver et renforcer. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis ce soir pour l’ultime étape de la longue navette entre votre hémicycle et celui

concrètement à la construction d’une véritable société du bien vieillir et de l’autonomie dans notre pays. J’aime cette expression de « bien vieillir », car elle fait écho à la formule du grand biologiste Étienne Émile Baulieu, qui a beaucoup fait progresser la recherche contre la maladie d’Alzheimer : « Vieillir n’est pas une maladie. Cette ambition du bien vieillir, je l’ai toujours faite mienne. Elle s’inscrit comme le fil rouge de l’action que mène le Gouvernement en la matière depuis 2017 et dont le Président de la République a toujours fait une priorité. effet, ce chantier, immense et essentiel, du grand âge s’achèvera non pas en un jour, mais au terme d’une action constante et résolue du Gouvernement et des parlementaires, avec les collectivités territoriales et toute la société. Je sais qu’il reste du travail, beaucoup de travail, et je suis pleinement mobilisée à vos côtés pour en venir à bout. C’est pourquoi le Gouvernement soutient ce texte pour ce qu’il est : une pierre supplémentaire d’un édifice plus large, apportant de nouvelles mesures utiles et concrètes à une action collective et de long terme qui se poursuit. Cette action résolue du Gouvernement s’est traduite entre autres par la création de la cinquième branche de la sécurité sociale, dédiée à l’autonomie, consacrée par la loi du 7 août 2020

Son budget, je veux le rappeler, s’élève à 40 milliards d’euros cette année et atteindra 45 milliards d’euros en 2027. Nous avons également lancé la réforme ambitieuse des services autonomie à domicile (SAD) en fusionnant le soin et l’aide à domicile, afin que chacun puisse être accompagné et soigné chez lui lorsqu’il le souhaite. Ce sont de véritables services intégrés qui mailleront ainsi tout le territoire, pour permettre au plus grand nombre de vieillir chez soi, en toute sécurité. Je pense aussi à la préfiguration du service public départemental de l’autonomie, porte d’entrée unique pour les personnes vieillissantes ou en situation de handicap, afin de les accompagner, de les orienter et de mieux prévenir la perte d’autonomie. Je souhaite qu’il soit généralisé dès 2025 ; grâce à cette proposition de loi, nous le préfigurons déjà dans 18 départements. Je tiens d’ailleurs à saluer ici l’engagement des départements préfigurateurs qui se sont portés volontaires. Je tiens également à mentionner le dispositif MaPrimeAdapt’, qui permet de financer, depuis le 1 janvier dernier, la réalisation des travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou en situation de handicap, en fonction de leurs besoins spécifiques. Il s’agit d’un dispositif très concret, qui accompagne ce virage domiciliaire indispensable, alors que 90 % des Français expriment le souhait de vieillir chez eux. Face à la crise de confiance qu’a pu connaître le secteur, nous avons mis en place le plan d’inspection générale des Ehpad, qui a déjà permis de contrôler la moitié des quelque 7 500 établissements pour personnes âgées du pays. J’ai annoncé lundi dernier, lors de la présentation de la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, que cette démarche d’inspection contrôle serait non seulement renforcée – l’objectif est d’avoir contrôlé 100 % des établissements avant la fin de l’année –, mais encore élargie aux établissements accueillant des personnes handicapées et systématisée, afin de l’inscrire dans la durée. Vous pouvez le constater, mesdames, messieurs les sénateurs, notre gouvernement a déjà fait beaucoup, avec vous, en faveur du grand âge. Avec vous, oui, car certaines des mesures figurant dans notre stratégie de lutte contre les maltraitances se trouvent également dans le texte que nous examinons aujourd’hui, permettant d’en assurer une effectivité rapide.

en mêlant exigence et ouverture au compromis, pour arriver à un texte efficace et respectueux de l’équilibre entre les différents acteurs du grand âge et de l’autonomie, notamment les collectivités départementales.

Je ne pourrai revenir sur l’ensemble des mesures de ce texte, mais je tiens à en citer quelques unes, particulièrement emblématiques de l’esprit de cette proposition de loi, qui met en place des changements concrets, ancrés dans la vie quotidienne, et qui répond à des besoins exprimés par les personnes et les acteurs du secteur.

Grâce à ce texte, on ne pourra plus, par principe, refuser à une personne âgée de recevoir son parent chez elle, car, oui, pour un résident, l’Ehpad est son lieu de vie, vie, son chez soi. Je souligne que ce droit inconditionnel de recevoir de la visite est aussi reconnu pour les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs. C’est dans le même esprit que je me réjouis de la place que nous donnons aux animaux de compagnie dans ces établissements. a confirmé la création d’un droit pour les résidents d’Ehpad d’accueillir leur animal domestique au sein des établissements, en prenant en compte la volonté du Sénat d’encadrer ce droit, afin de garantir la santé et la sécurité des résidents et du personnel, ainsi que le bien être des animaux. C’est pourquoi je prends devant vous l’engagement de travailler à un décret d’application équilibré, rédigé après concertation avec les professionnels et les associations, afin que ce droit s’applique dans le respect le plus strict des exigences d’hygiène et de sécurité.

Je pourrais aussi mentionner le renforcement de l’habitat inclusif ou encore les dispositions concernant la lutte contre les maltraitances, dont certaines font partie de notre stratégie nationale,

Pour reprendre une formule de M. Mouiller,… De l’excellent M. Mouiller ! … ce texte « aborde des questions qui se posent avec une intensité croissante avec le vieillissement de la population, sans toutefois les épuiser

évidemment pas la question centrale du financement, afin de décider collectivement qui paie quoi, entre la sécurité sociale et l’État, entre les différentes générations,

C’est pourquoi je m’engage ici à ce que nous en débattions avec vous, avec tous les Français, afin de tirer toutes les conséquences nécessaires, y compris, bien entendu, dans la loi. Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi est un pas de plus dans la mise en œuvre d’un modèle social renouvelé, pour une meilleure prise en charge de la dépendance.

dans le quotidien de ceux qu’elles visent. Humaniser les établissements, renforcer le domicile, lutter contre les maltraitances, tout cela est bel et bien

mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, grâce aux progrès de la médecine et à l’amélioration des conditions de vie, la France est confrontée à d’importants changements démographiques : ceux qui ont grandi pendant les Trente Glorieuses arrivent massivement à l’âge où beaucoup deviennent dépendants. Si l’espérance de vie progresse, cet âge correspond malheureusement trop souvent à des mois passés en mauvaise santé. Selon les estimations du rapport Libault, entre 2,7 et 3,7 millions de personnes deviendront dépendantes dans les années à venir. Ce mur de la dépendance nous impose de mettre en place une véritable politique pour répondre aux défis du vieillissement de la population. Maintes fois promis et maintes fois reporté, ce chantier hante les gouvernements successifs depuis plus de vingt ans. Grâce à l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, cette réforme devrait prendre la forme d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge, la première, qui devrait être présentée avant la fin de l’année. Certes, comme l’a rappelé le président du conseil de la CNSA, ce n’est pas tout à fait la grande réforme que nous attendions. que nous attendions. Mais cela s’en approche. Votre prédécesseur l’avait affirmé, madame la ministre, devant l’Assemblée nationale : « La loi de programmation que vous, parlementaires, avez demandée […] constitue une fondation essentielle. […] [L]’arbitrage a été rendu, l’engagement est pris. »

Dans cette attente, la proposition de loi que nous nous apprêtons à voter constitue une première étape. Elle comporte des mesures importantes, et les débats, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, ont permis de l’enrichir. Je remercie les deux rapporteurs ici présents de leurs travaux fructueux. Nous saluons Nous saluons ainsi la création d’un service public départemental de l’autonomie (SPDA), qui permettra aux personnes âgées ou en situation de handicap et à leurs aidants d’avoir facilement accès à l’information et d’être efficacement orientées en fonction des besoins.

renforce le rôle du département comme chef de file des politiques de soutien à l’autonomie, tout en tenant compte des spécificités de certains territoires. C’est une très bonne chose. En matière de prévention de la perte d’autonomie, plusieurs mesures méritent d’être soulignées. Nous saluons également le versement d’une aide financière annuelle aux départements pour soutenir les aides à la mobilité des intervenants à domicile. Cette aide est d’autant plus précieuse que les déplacements représentent une contrainte majeure, qui nuit à l’attractivité d’un métier pourtant essentiel.

un mot de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, qu’elle soit organisée, comme l’a révélé le scandale Orpea, ou institutionnelle, par manque de moyens et de personnel. Comme l’a rappelé la Défenseure des droits, 281 réclamations ont été reçues entre mai 2021 et janvier 2023, confirmant, « le caractère systémique du problème de maltraitance au sein des Ehpad ». Nous saluons la mise en place d’une cellule de recueil et de traitement des alertes à l’échelon du département, ainsi que l’élargissement des compétences de la Conférence nationale de santé (CNS) à la question de la lutte contre la maltraitance. Faisant écho au rapport intitulé de novembre dernier, le texte consacre enfin un droit de visite pour les résidents en Ehpad, les personnes hospitalisées et les personnes en fin de vie, pour que les situations inhumaines qui ont eu lieu pendant l’épidémie de covid ne puissent plus jamais se reproduire. Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE apportera son soutien à cette proposition de loi, conscient toutefois qu’elle n’est pas la grande loi tant attendue. une loi qui assurera une meilleure collaboration entre tous les acteurs de la prise en charge de l’autonomie, une loi qui garantira une gouvernance claire et lisible pour l’usager, une loi qui assurera une source de financement fiable, juste et pérenne pour les conseils départementaux, une loi, enfin, qui permettra

la prise en charge du vieillissement de la population, tout en garantissant une vie de qualité et un cadre de vie décent pour tous. Tel est l’objet de la présente proposition de loi, et je souhaiterais tout d’abord rendre hommage aux députées de la majorité présidentielle qui en sont à l’origine : les rapporteures, Mmes Laurence Cristol et Annie Vidal, ainsi que

ensuite, combattre les maltraitances des personnes en situation de vulnérabilité et garantir leurs droits fondamentaux ; enfin, garantir à chacun des conditions d’habitat dignes, ainsi que des prestations de qualité et accessibles, grâce à des professionnels accompagnés et soutenus dans leurs pratiques. Je me réjouis que le compromis issu de la commission mixte paritaire préserve l’équilibre du texte que nous avions voté au Sénat. Différents amendements du groupe RDPI adoptés ici ont été repris dans le texte issu de la comme sur le service public départemental de l’autonomie : face aux difficultés de pilotage des politiques de l’autonomie, ce service sera le lieu de la coordination et de la planification pluriannuelle Je souhaiterais aussi rappeler mon amendement sur la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins dans les aides à la mobilité, pour faire face aux difficultés de continuité territoriale et ainsi contribuer à redonner de l’attractivité au métier d’aide à domicile sur l’ensemble du territoire national. Le texte issu de la commission mixte paritaire conserve par ailleurs le caractère inconditionnel du droit de recevoir de la visite en établissement, pour les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs. Nous nous réjouissons enfin des compromis trouvés sur la transformation des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) en services autonomie à domicile (SAD), sur la tarification de l’hébergement en Ehpad, ou encore sur la création d’un droit, pour les résidents en Ehpad, de voir leur animal domestique accueilli accueilli au sein des établissements. Vous le voyez, mes chers collègues, cette proposition de loi comporte de nombreuses mesures qui vont dans le sens d’une meilleure prise en charge du vieillissement et d’une amélioration de la politique de l’autonomie. Ce texte n’est peut être qu’une brique, mais celle ci est utile dans nos efforts pour prendre en charge le vieillissement et garantir une vie de qualité à nos aînés, dans un cadre de vie décent. Nous voterons donc pour, sans hésitation. Madame la ministre, avec cette proposition de loi, les parlementaires ont pris leurs responsabilités. Nous attendons maintenant que le Gouvernement fasse de même, en nous proposant une loi sur le grand âge Malgré la situation budgétaire délicate, il faut se retrousser les manches et travailler à des solutions innovantes, par exemple sur le sujet de la gouvernance ou encore sur le financement de la politique de l’autonomie. Nous devrons également continuer à agir pour redonner de l’attractivité au secteur, qui en manque cruellement depuis des années, et enfin continuer à être vigilants sur le contrôle des Ehpad, pour que les scandales récents ne se reproduisent plus. À ce titre, la mission de contrôle sur la situation des Ehpad, dont je suis corapporteure, rendra ses conclusions à la fin du semestre. Enfin, madame la ministre, comment conclure sans dire un mot sur l’outre mer Face à un vieillissement de la population encore plus fort et à un parc des Ehpad très vieillissant, il nous faudra des réponses rapides pour que le bien vieillir soit une réalité partout, dans l’Hexagone comme en outre mer.

de nos proches ; nous sommes toutes et tous concernés. Nous devons faire face à un véritable défi démographique, social et humain. Le vieillissement de la société requiert une vision panoramique et des actions d’ampleur dans un grand nombre de domaines. Or cette proposition de loi ne constitue qu’un patchwork de mesures, souvent vagues et bien insuffisantes. Pour dépasser l’invisibilisation de nos aînés et de ceux qui les accompagnent, aidants familiaux et professionnels, une planification méthodique et le vote de moyens dédiés s’imposent. Gardons tous à l’esprit que le vieillissement ne signifie pas la fin de la vie. Les personnes âgées ont besoin d’un accompagnement adapté, qui fait souvent défaut aujourd’hui. Oui, les attentes de nos concitoyens et des professionnels du secteur du grand âge sont légitimement fortes. Il est impératif d’y répondre, non pas par une simple proposition de loi, mais bien par un projet de loi de programmation d’ampleur, comprenant une véritable trajectoire financière. Ce dont ont besoin les personnes vieillissantes et les professionnels qui en prennent soin, ce n’est pas de « diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie » comme le suggère le titre de cette Ils ont besoin que le Gouvernement honore les engagements pris, que la grande loi sur le grand âge, promise par le Président Emmanuel Macron il y a six ans – bientôt sept ! – soit enfin discutée et votée. Sans cesse ajournée, elle ne figure pas parmi les textes dont le Gouvernement prévoit l’inscription à l’ordre du jour prioritaire jusqu’à la fin de la session ordinaire. Faut il définitivement en conclure, madame la ministre, que ce gouvernement ne présentera aucun texte d’ampleur sur le grand âge ? Nous attendons une réponse claire. Depuis plusieurs semaines, nous regrettons que le Gouvernement se mure dans le silence. Il nous paraît inconcevable et surtout irresponsable que le Premier ministre Gabriel Attal ne reprenne pas l’engagement clair de sa prédécesseure, Mme Élisabeth Borne, qui s’était engagée à faire adopter une vraie loi Grand Âge d’ici à la fin de l’année c’est à dire aujourd’hui ! Nous appelons donc le Premier ministre à confirmer les engagements pris devant la représentation nationale, et vous, madame la ministre, à lancer rapidement un travail de coconstruction avec les acteurs du secteur, que Mme Aurore Bergé, alors ministre des solidarités et des familles, avait évoqué.

Que leur répondez vous ? Là encore, sans réponse de votre part, madame la ministre, parler du bien vieillir n’a aucun sens. Qu’en est il du droit à vieillir dignement ? Il est nécessaire de donner une suite législative à cette proposition, qui ne peut en aucun cas se limiter au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) de l’automne prochain. C’est une loi de programmation pluriannuelle, sur cinq ans, dont nous avons besoin. Malgré toutes vos promesses, vous n’arrivez même pas à mobiliser les moyens humains nécessaires pour accompagner le grand âge à domicile ou dans les établissements dédiés.

repoussé l’échéance, en évoquant désormais l’horizon de l’année 2030. Ces recrutements sont précisément l’enjeu d’une loi de programmation, avec des financements associés. Il n’est pas sérieux de multiplier ainsi les promesses non tenues et de repousser continuellement des mesures vitales pour tant de nos concitoyens. Logiquement, les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ont donc décidé de s’abstenir sur ce texte, tristement conscients que tout

Le texte consacre certaines avancées : le service public départemental de l’autonomie, avec notamment la possibilité de définir des territoires de l’autonomie à l’échelon infradépartemental ; la généralisation du programme Icope en matière de prévention l’inscription du droit de visite inconditionnel en Ehpad et pour les personnes en fin de vie ou en soins palliatifs ; la création, au 31 décembre 2026, d’un registre général des mesures de protection juridique, regroupant les mesures judiciaires et les mandats de protection future l’instauration d’une carte professionnelle pour les personnels du secteur du domicile après trois années d’exercice professionnel ; la possibilité donnée aux Ehpad habilités à l’aide sociale de moduler leurs tarifs

J’en viens à la réforme qui prévoit le regroupement de l’ensemble des services à domicile existants en une unique catégorie dénommée services autonomie à domicile. Depuis

d’une part, elle leur a donné un délai supplémentaire de six mois pour déposer une demande d’autorisation en SAD, reportant l’échéance au 31 décembre 2025 d’autre part, elle a prévu l’extension de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle un Ssiad peut conclure une convention ou former un groupement avec un service proposant des prestations d’aide et d’accompagnement, à défaut de présenter une demande d’autorisation. Madame la ministre, nous ne sommes pas opposés à cette réforme, mais force est de constater que sa mise en place est chaotique. Il est donc indispensable de bien accompagner les Ssiad, pour ne pas mettre en péril leur intervention auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. dressée la liste de ces mesures, nous pouvons affirmer qu’elles ne constituent qu’une réponse partielle aux enjeux du vieillissement de la population. Nous attendons désormais l’examen d’un projet de loi, d’une loi cadre ou d’une loi de programmation – les termes ne sont pas importants ce qui est essentiel, c’est de débattre, rapidement, pour affecter de nouveaux moyens financiers à la branche autonomie. À l’heure où une large majorité d’Ehpad connaît de graves difficultés financières

Les 100 millions d’euros alloués à ce titre l’an dernier sont d’ores et déjà consommés. Ce ne sont pas de crédits d’urgence que les acteurs de l’autonomie ont besoin, mais bien de financements pérennes. De plus, le virage domiciliaire ne peut rester qu’un slogan.

Il est donc urgent de rassurer l’ensemble des directeurs d’établissement et l’ensemble des structures intervenant à domicile, et de répondre aux attentes de nos concitoyens. Madame la ministre, quel calendrier

Comme souvent en Macronie, nous ne pouvons qu’adhérer aux annonces, mais les actions et les faits sont toujours têtus. Un tel texte aurait dû conduire à un consensus, s’il avait été construit dans un esprit d’écoute et de travail en commun. composé d’une quinzaine d’articles lors de son dépôt, les parlementaires ont intégré une cinquantaine d’articles additionnels. Ces différents ajouts montrent une appétence de la représentation nationale pour ce sujet, qui est un enjeu essentiel pour notre vie en société. Comme souvent en Macronie, on fait des promesses. Le Président de la République avait annoncé en 2018 une grande loi pour répondre aux défis du vieillissement… À quand la loi Grand Âge, ambitieuse, nécessaire, attendue, tant promise ? Comme souvent en Macronie, ce texte manque d’une vision globale. Le Gouvernement n’a pas su s’emparer d’un sujet si important et qui soulève, au delà d’enjeux concrets et pragmatiques, un enjeu moral. Comment voulons nous écouter, accompagner et soutenir nos aînés, qui sont le maillon fort de notre société et ont souvent contribué à sa richesse, qui sont porteurs des valeurs que nous défendons, comme la famille et le travail ? Ils méritent une reconnaissance nationale par un accompagnement digne et humaniste pendant ce chapitre qui conclut leur parcours de vie. La commission des affaires sociales du Sénat, dans sa sagesse, a bien souligné que la proposition de loi n’entraînera pas de bouleversement des politiques de soutien à l’autonomie. Après un travail de mise en commun et de discussions constructives pendant la commission mixte paritaire, quelques mesures pertinentes sont ressorties et vont dans le bon sens. En effet, la sanctuarisation du droit de visite est une belle avancée. Rappelons que, pendant la crise de la covid, nombre de nos concitoyens ont conclu leur vie sans pouvoir être accompagnés par leurs proches, un traumatisme que notre société ne doit plus jamais subir. à la suppression de l’article 1 , qui permet de maintenir l’avis du maire sur la nomination des directeurs d’Ehpad. Rappelons ici que les maires connaissent leur territoire et leurs concitoyens. Il est donc essentiel et légitime qu’ils puissent avoir un droit de regard et de parole lors d’une telle décision. Le Rassemblement national souhaite, comme d’autres partis politiques, qu’un véritable projet de loi soit proposé à la représentation nationale, avec une mise en avant des professionnels du secteur, non pas avec une carte professionnelle, relevant plutôt du symbole, mais avec un réel statut, une réelle formation continue et une rémunération digne avec une reconnaissance du proche aidant dans le processus de soins et de maintien à domicile ; avec une réforme des Ehpad ou une remise à plat des fonctionnements et des financements. En effet, force est de le constater, face aux situations financières difficiles de nombreux établissements, face à l’épuisement des professionnels, l’épuisement des professionnels, face aux actes de maltraitance qui se multiplient, l’Ehpad d’aujourd’hui ne répond plus de manière efficiente aux enjeux qui lui sont imposés, malgré une volonté sans faille du secteur. Nous devons collectivement remettre l’humain au centre de tous les défis. défis. Même si cette proposition de loi n’est pas la grande loi tant attendue, tant promise, elle apporte de petites avancées. Nous votons donc pour ce texte. La parole est à Mme Corinne Bourcier, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

quasiment un an, c’est long… C’est le temps qu’il aura fallu à cette proposition de loi pour être examinée par le Parlement, depuis les premières séances à l’Assemblée nationale jusqu’à aujourd’hui.

Nous sommes satisfaits du maintien de la plupart des choix de notre chambre dans la version finale du texte, même si ce dernier ne provoquera pas de grand chambardement dans le domaine du grand âge – telle n’était pas non plus sa prétention. Pour ma Pour ma part, je me réjouis du rétablissement de la conférence nationale de l’autonomie. Je pense que cela permettra de mettre ce sujet au centre des préoccupations, c’est à dire au niveau qu’il mérite. La mise en place du fameux service départemental de l’autonomie est une évidence pour faciliter la coordination des acteurs et rendre plus simple et efficace le parcours des personnes âgées en situation de handicap et de leurs proches. Les établissements pourront désormais utiliser leur forfait soins pour mener des actions de prévention contre la dépendance. Cela paraît évident et, pourtant, ils n’étaient jusqu’à maintenant pas autorisés à le faire. Au delà de son aspect pratique dans le budget des établissements, je me réjouis de cette mesure, car elle démontre une évolution dans la façon de considérer ce qu’est le soin : en quelque sorte, elle reconnaît que la prévention est du soin à part entière.

qui, comme je l’avais proposé, a été étendue à tous les professionnels intervenant à domicile. Il s’agira d’avancées très concrètes pour les professionnels concernés. Par ailleurs, je suis largement favorable à ce qu’un Ehpad puisse accueillir un animal de compagnie, de façon permanente ou lors d’activités de médiation animale. Les bienfaits des animaux sont connus et reconnus. la vie en Ehpad est une vie en collectivité. Je reste convaincue que promettre aux personnes âgées qu’elles pourront garder leur animal de compagnie en entrant en Ehpad est une fausse promesse, car une telle mesure sera inapplicable sur le terrain. Le texte contient enfin quelques mesures pour lutter contre la maltraitance, comme la création d’une cellule départementale dédiée aux signalements ou encore la garantie d’un droit de visite pour les personnes accueillies en établissement. J’avais eu l’occasion de le dire lors des explications de vote sur ce texte, en première lecture : selon moi, le meilleur moyen de lutter contre la maltraitance, c’est d’avoir du personnel en nombre suffisant, correctement formé et rémunéré. Cela ne veut pas dire que d’autres mesures ne sont pas importantes pour lutter contre la maltraitance, mais le personnel reste la condition préalable et indispensable. Pour les quelques améliorations concrètes que ce texte propose et que notre groupe souhaite soutenir, nous voterons pour cette proposition de loi. il est vrai que le texte n’apporte pas de nouvelles perspectives financières. Or celles ci sont indispensables si nous voulons que nos aînés soient dignement traités en établissement, et si nous voulons réussir le virage domiciliaire domiciliaire et respecter ainsi le souhait des 85 % de Français qui veulent vieillir chez eux. Madame la ministre, nous attendons donc toujours un projet de loi, avec des orientations chiffrées, comme l’a promis Mme la ministre Vautrin devant notre commission.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte, dont j’ai eu l’honneur d’être rapporteure aux côtés de M. Jean Sol, n’est peut être pas la grande loi attendue sur le grand âge et l’autonomie, mais il nous permet d’avancer sur des sujets de préoccupation pour les Français. Je concentrerai mon propos sur les dispositions que j’ai plus particulièrement suivies en tant que rapporteure. Tout d’abord, le texte de la commission mixte paritaire consacre le droit du patient ou du résident de recevoir de la visite, en maintenant le régime proposé par le Sénat pour les établissements de santé et les établissements médico sociaux. Le texte inscrit dans la loi le droit inconditionnel, même en cas de crise sanitaire, reconnu aux personnes en fin de vie ou en soins palliatifs de recevoir de la visite, tout en précisant que l’établissement doit garantir les consignes de protection sanitaire. En outre, il étend ce droit inconditionnel à tout visiteur choisi par le patient ou résident et, si son consentement ne peut être exprimé, à tout membre de sa famille, de ses proches ou à la personne de confiance désignée. À l’article 4, qui prévoit un nouveau circuit de recueil et de traitement des cas de maltraitance commis sur des majeurs vulnérables, la commission mixte paritaire a adopté une rédaction de compromis prévoyant une cellule de recueil et de suivi des signalements pilotée par l’agence régionale de santé, selon la configuration prévue par l’Assemblée nationale. Ce dispositif s’accompagnera du déploiement d’un nouveau système d’information mis en œuvre par l’État. En revanche, deux apports du Sénat sont maintenus. D’une part, le numéro national d’appel, le 39 77, conserverait une base légale. D’autre part, le signalement des cas de maltraitance par les personnes astreintes au secret professionnel resterait une faculté, qu’ils apprécieraient en conscience. En matière de contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, le texte de la commission mixte paritaire entérine la rédaction adoptée par le Sénat. Le texte étend toutefois le périmètre de l’attestation transmise à l’employeur aux condamnations non définitives et aux mises en examen dont est frappé, le cas échéant, le professionnel ou la personne bénévole concernée. Enfin, nous nous sommes entendus pour maintenir la suppression de la plupart des articles relatifs à la protection des majeurs, suivant en cela l’avis de notre collègue Elsa Schalck, au nom de la commission des lois. J’en viens à la partie du texte concernant les services à domicile. Les deux assemblées ont approuvé la création d’une carte professionnelle pour les intervenants à domicile. La majorité d’entre eux ne disposant d’aucun titre ou diplôme, le Sénat a prévu d’autoriser la délivrance de cette carte aux personnes justifiant de deux années d’exercice professionnel. Par cohérence avec le cahier des charges des autorisations et des agréments, la CMP a rehaussé cette condition d’ancienneté à trois ans. Comme l’avait souhaité le Sénat, une partie de la contribution de la CNSA aux départements au titre de la mobilité des aides à domicile pourra être affectée à des aides financières à l’obtention du permis de conduire, sous réserve que les professionnels ne puissent bénéficier d’aucun autre dispositif visant le même objectif. Le regroupement des catégories existantes de services à domicile en une unique catégorie dénommée « services autonomie à domicile » implique une transformation qui se révèle difficile en pratique, notamment pour les services de soins infirmiers à domicile ; ceux ci disposent d’un délai de deux ans pour s’adjoindre une activité d’aide, fusionner ou se regrouper avec un SAD existant. L’article 8 vise à répondre à ces difficultés et aux inquiétudes qu’elles suscitent en permettant aux Ssiad de conventionner avec un SAD pendant une durée de trois ans sans demander de nouvelle autorisation. Il prévoit, en outre, un délai supplémentaire pour les Ssiad essuyant un refus d’autorisation, que le Sénat a fixé à deux ans. ans. Le Sénat avait également adopté un article 8 ayant pour objectif de rendre facultative l’application de la réforme par les Ssiad. Après de longues discussions sur ce sujet complexe, nous avons estimé que la mise en œuvre de cette réforme, que nous avons votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, est désormais trop avancée pour permettre tout retour en arrière. En contrepartie de la suppression de l’article 8 , la CMP a introduit à l’article 8 des assouplissements supplémentaires en faveur des Ssiad la durée pendant laquelle ils pourront se maintenir dans le cadre d’une convention ou d’un groupement, à défaut de présenter une demande d’autorisation en SAD, est allongée à cinq ans, et la date butoir pour déposer cette demande d’autorisation est repoussée de six mois, soit au 31 décembre 2025. Ce compromis, doublé d’un engagement du Gouvernement de mieux accompagner les Ssiad dans cette transformation, me semble de nature à sécuriser le sort de ces services. L’article 10 permettra aux Ehpad majoritairement habilités à l’aide sociale de fixer des tarifs différenciés entre les personnes bénéficiaires de l’aide sociale et les autres, dans la limite d’un écart fixé au niveau national par décret et à condition de maintenir une part suffisante de bénéficiaires de l’aide sociale parmi les résidents. Les départements auront toujours la possibilité de fixer des conditions plus strictes que le cadre national. Je me réjouis enfin que nous soyons parvenus à trouver un accord sur la base du texte adopté par le Sénat pour ce qui concerne les articles dédiés à l’habitat inclusif et aux résidences autonomie. Mes chers collègues, je vous invite

collègues, le journal résumait parfaitement ce matin les enjeux du texte qui nous réunit : « Un dernier vote au Sénat qui peinera à masquer les inquiétudes des parlementaires sur l’avenir du secteur de l’autonomie, en l’absence de promesse gouvernementale pour une prochaine loi sur le grand âge.

rien. Quand le Gouvernement promet au Parlement la présentation d’un projet de loi sur le grand âge au premier semestre, mais que rien n’est inscrit à l’ordre du jour

Ce texte comporte des propositions intéressantes : droit sanctuarisé de visite dans les Ehpad, possibilité d’accueillir des animaux en établissement, instauration d’un droit de visite pour les proches, création d’une carte professionnelle pour les aidants.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est donc parvenue à un accord au rabais, sur un texte sans envergure, dont le financement est insignifiant. Cette proposition de loi comporte certes quelques mesures positives, comme la dotation de 100 millions d’euros pour aider les départements à financer la mobilité des intervenants à domicile. la sanctuarisation d’un droit de visite pour les résidents des Ehpad et à la possibilité d’accueillir un animal de compagnie. Toutefois, ces dispositions sont bien loin de compenser les reculs et les manques de ce texte. La commission mixte paritaire a supprimé de cette proposition de loi l’obligation de réserver une part des bénéfices des Ehpad privés lucratifs à l’amélioration des conditions de vie. Elle a également supprimé l’obligation faite de se conformer aux injonctions de l’ARS en cas de constatation de manquements graves à la qualité et à la sécurité des soins. Malgré l’ampleur des révélations du livre, vous vous préférez protéger les directions des Ehpad maltraitants, plutôt que les résidents. Alors que le Président de la République avait annoncé la création de 50 000 postes, seulement 3 000 ont été ouverts en 2023 et 6 000 en 2024. L’objectif de 50 000 postes a donc été repoussé de 2027 à 2030, alors même que les besoins sont estimés par l’association des directeurs d’Ehpad à 200 000 emplois supplémentaires. Tant que les gouvernants refuseront d’investir dans le secteur médico social, le personnel continuera de subir la maltraitance institutionnelle et les résidents des conditions dégradées de prise en charge. a pourtant urgence : selon la Fédération hospitalière de France, le nombre d’Ehpad en déficit est passé de 45 % à 85 à 85 % entre 2019 et 2022 et le coût unitaire d’un lit a bondi de presque 10 %, pour atteindre un déficit unitaire moyen de 3 200 euros.

Nous connaissons les ordres de grandeur que suppose un tel projet : il faudrait 10 milliards d’euros, soit l’équivalent du plan d’austérité de Bruno Le Maire pour 2024. Nous avons quelque peine à croire que le Gouvernement, qui annonce 30 milliards d’euros d’économies l’an prochain et qui souhaite réduire les dépenses des personnes en affection de longue durée, propose une loi de programmation de financement du secteur du grand âge et de l’autonomie… Depuis 2017, nous sommes dans l’attente impatiente d’une loi sur le grand âge pour financer l’adaptation de la société au vieillissement. Il suffirait pourtant de mettre à contribution les plus hauts revenus et les revenus financiers ou de revenir sur les 88 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales

sur la revalorisation des métiers de l’aide à domicile, rien sur la revalorisation des salaires des personnels, rien sur la revalorisation des frais kilométriques des aides à domicile qui utilisent leur véhicule personnel Ce n’est pas en appliquant les méthodes du secteur privé lucratif que nous allons améliorer la situation des Ehpad publics et privés non lucratifs tarifs différenciés selon les revenus des résidents ne va pas améliorer le taux d’encadrement ni la qualité de l’accueil ; au contraire, cela risque de réduire encore le nombre des places réservées à l’aide sociale. L’affaire Orpea a pourtant mis en lumière les dysfonctionnements du secteur privé lucratif, avec des montages financiers ayant pour seul objectif la recherche d’une rentabilité maximale, au mépris des êtres humains.